Ma question s'adresse à Mme la Première ministre. Le prince-président nous a gratifiés à l'heure méridienne de sa bonne parole. Totalement hors-sol, il a annoncé continuer à avancer à marche forcée. Totalement hors-sol, il a osé comparer l'un des plus grands mouvements populaires de notre histoire à la sédition factieuse des suprémacistes blancs envahissant le Capitole. Totalement hors-sol, il a insulté les manifestantes et les manifestants, sans avoir un mot pour condamner les exactions de la police, qui, sous vos ordres, tabasse, nasse, jette des grenades en pleine tête, roule à moto sur les gens, intimide et arrête n'importe qui, n'importe quand, sous le regard alarmé du Défenseur des droits. Totalement hors-sol et plus à une incohérence près, il a tout de même reconnu que cette réforme était brutale et, surtout, qu'elle ne s'intéressait ni à la réalité du travail, ni à la pénibilité, ni aux fins de carrière, ni aux reconversions. Madame la Première ministre, avec gravité, avec inquiétude, nous vous le demandons solennellement : revenez à la réalité et retirez cette réforme avant d'avoir un drame sur la conscience.

Oui, cette réforme est nécessaire pour assurer l'avenir de nos retraites. N'importe quoi ! Sans elle, les déficits s'accumuleraient et nous serions contraints à des hausses d'impôts ou à des baisses de pensions, au détriment des plus modestes et des classes moyennes.

Oui, le compromis fonctionne. Nous avons travaillé ensemble, bâti un projet qui reprend des propositions que la majorité sénatoriale prônait parfois depuis longtemps, mais aussi des idées qui n'étaient pas les vôtres, issues de l'Assemblée Ce projet, vous l'avez adopté par deux fois à une large majorité. C'est la méthode Coué ! À cet égard, je tiens à saluer les membres de la majorité sénatoriale et ceux qui soutiennent l'action du Président de la République pour leur engagement au service de notre modèle social. Enfin, oui, nous avons respecté l'esprit et la lettre de la Constitution et nous sommes arrivés au terme du cheminement parlementaire de cette réforme. En revanche, non, on ne peut pas brader l'intérêt général par démagogie ou par peur de l'impopularité. Non, les violences ne sont pas excusables et je veux rendre hommage à nos policiers et à nos gendarmes pour leur engagement au service de l'ordre républicain.

Je pense à cette demande de justice : nous devons veiller à ce que les travailleurs bénéficient davantage des profits exceptionnels de certaines entreprises. En taxant les superprofits ? Je pense aux attentes de nos concitoyens dans leur rapport au travail, à notre capacité à prévenir l'usure professionnelle et à offrir des perspectives de carrière à chacun. En les faisant travailler deux ans de plus ? Nous devons continuer sur le chemin de la réindustrialisation et du plein emploi, car ils permettront d'assurer notre souveraineté et l'avenir de notre modèle social. Nous devons veiller à l'ordre républicain en prévoyant des moyens supplémentaires pour nos forces de l'ordre et notre justice. Nous devons permettre à nos compatriotes de vivre mieux en prenant des décisions aux effets sensibles et rapides, en travaillant avec nos collectivités sur la santé, sur l'éducation et sur la transition écologique. Ce cap fixé, le Président de la République m'a chargée d'engager un travail avec tous les parlementaires qui veulent agir pour notre pays. Nous en sommes capables, nous l'avons montré encore récemment en bâtissant des majorités de projet,

Même les ressorts autoritaires de nos Constitutions d'un autre temps sont brisés. Vous ne pouvez pas gouverner en technocrate de palais contre le peuple. Nous sommes entrés cette semaine dans un de ces moments récurrents de notre histoire où le fleuve de la colère populaire est sorti de son lit. Seul le pouvoir exécutif peut en tarir la source et rétablir le calme. Retirez votre réforme et remettez tout à plat- le travail, la retraite -, comme l'a lui-même annoncé le Président de la République tout à l'heure. Tant que vous y êtes, lancez aussi la refonte de nos institutions anachroniques pour que les mots du Président de la République- « J'ai le sens de la démocratie. » -ne soient pas un énième mensonge, une énième provocation. Vous n'avez de toute façon plus de majorité pour faire autre chose.

Dans un contexte de forte inflation, nos entrepreneurs sont préoccupés. Ils ont suivi avec beaucoup d'attention les incidents des secteurs bancaires étrangers, ainsi que les réponses apportées par les régulateurs. Indispensable pour contenir l'envolée des prix, qui ronge le pouvoir d'achat de nos concitoyens, la hausse des taux directeurs entraîne dans le même temps un renchérissement du crédit. Alors que l'investissement est toujours nécessaire à une économie en croissance, il l'est encore davantage lorsque l'on a pour ambition de réindustrialiser le pays. Le Président de la République a rappelé à plusieurs reprises combien il était essentiel à notre souveraineté que nous puissions de nouveau produire en France.

Aujourd'hui, le chef de l'État a annoncé la mise en place prochaine d'une contribution des entreprises en faveur des salariés. Monsieur le ministre, dans un contexte où nos entreprises ont autant besoin d'être rassurées que nos concitoyens, pourriez-vous nous donner des éclaircissements sur ce nouveau dispositif ? S'agit-il d'une nouvelle taxe ? Comment la compétitivité et la capacité d'investissement de nos entreprises seront-elles préservées ?

de la souveraineté industrielle et numérique. Madame la sénatrice Colette Mélot, nous partageons totalement votre objectif de trouver le bon équilibre entre la compétitivité des entreprises, notamment de notre industrie, et la nécessité de mieux partager la valeur pour les salariés, pour que tous ceux qui travaillent en aient tout simplement pour leur engagement. C'est ce que nous avons fait depuis six ans. Nous avons simplifié l'intéressement et les accords de participation. Nous avons supprimé la taxe à 20 qui pesait sur les accords d'intéressement et de participation. Nous avons mis en place, en accord avec le Président de la République, la prime défiscalisée jusqu'à 6 000 euros pour redistribuer de la valeur aux salariés. Nous avons également demandé à toutes les entreprises qui bénéficient de rentes- je pense aux entreprises énergéticiennes -de redistribuer cette rente par le biais de la contribution sur la rente inframarginale, qui rapporte plusieurs milliards d'euros et qui finance le bouclier énergétique que nous avons mis en place avec la Première ministre. La proposition du Président de la République est la troisième étape de cette meilleure répartition de la valeur entre le salarié et l'entreprise. Nous voulons que les entreprises qui font du rachat d'actions contribuent davantage à une meilleure rémunération des salariés, Nous voulons les obliger à distribuer plus d'intéressement, plus de participation, plus de primes défiscalisées, lorsqu'elles font du rachat d'actions. Nous voulons que ce soit substantiel. Nous pourrions par exemple envisager un doublement des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ou des primes défiscalisées pour toutes les grandes entreprises qui font du rachat d'actions. De quelles entreprises parlons-nous ? Nous parlons des grandes entreprises, celles qui comptent plus de 5 000 salariés et celles qui font

je vous remercie de nous avoir rappelé les mesures qui avaient déjà été prises et les nouvelles mesures dont nous attendons, bien sûr, nombreuses retombées- une nouvelle répartition, une contribution des grandes entreprises -, afin que l'intéressement et la participation puissent

Sa réponse s'était alors voulue rassurante : le dispositif serait corrigé « dans les toutes prochaines semaines », une échéance ayant été fixée au « début du mois de mars, pas plus tard » ! Depuis, cette échéance est sans cesse repoussée.

En dépit de solutions temporaires telles que la réouverture d'Infogreffe, ce service de simplification continue de dysfonctionner jusqu'à compromettre en particulier l'avenir de la filière artisanale. Première difficulté, le registre national des entreprises n'est pas fiable et ne comporte aucune mention d'appartenance au secteur des métiers et de la qualité artisanale. Les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) sont dans l'incapacité de fournir des extraits d'inscription issus du registre national, la synthèse obtenue après validation n'étant pas reconnue par les partenaires, banques et assureurs. Seconde difficulté, la complexité du système de catégorisation est telle que les entreprises artisanales ne sont tout bonnement plus identifiées L'alerte est donnée, les chambres des métiers et de l'artisanat ne peuvent plus exercer leurs missions de contrôle. Elles sont contraintes de maintenir leurs logiciels métiers en doublon du guichet unique, ce qui représente un coût important. Le réseau des CMA a formulé des propositions. Madame la ministre, quelles suites allez-vous y donner ? Quelles mesures allez-vous prendre pour fiabiliser le registre issu du guichet unique et permettre une meilleure identification de l'activité et de la qualification artisanales ? je vous remercie

Je pense au problème des multi-validations qui se pose quand un artisan doit obtenir la validation de ses données non seulement par la CMA, mais aussi par le greffier du tribunal de commerce. Mes services se sont saisis du sujet, ils accélèrent leurs travaux pour améliorer et faciliter le partage d'informations. La qualité et la précision du registre national des entreprises sont aussi un enjeu. Ce registre, que vous connaissez, a été conçu pour regrouper les données de toutes les entreprises. Il est légitime que les entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat soient clairement identifiées en tant que telles au sein du registre. Des insuffisances demeurent encore

Ce document, très attendu, résonne comme un coup de semonce. L'humanité est au pied du mur. Face au réchauffement climatique, c'est agir ou périr. Monsieur le ministre, le gouvernement auquel vous appartenez et l'Union européenne en ont bien conscience, ce dont témoignent les efforts d'accélération de la transition environnementale.

un service qui dépend de Matignon et dont la qualité des travaux n'est plus à démontrer, la transition écologique pourrait avoir le même effet que la désindustrialisation ayant eu lieu depuis 1997. À l'heure où Bercy achève la coconstruction de son projet de loi pour une industrie verte, le problème est crucial. Les auteurs de l'étude soulignent que, « selon la Commission européenne, entre 35 % et 40 % des emplois pourraient être touchés par la transition écologique La question clé est de savoir s'il pourra y avoir une réallocation de main-d'oeuvre fluide entre les secteurs gagnants, c'est-à-dire les secteurs décarbonés, et les secteurs polluants. Dans la situation actuelle, rien n'est moins sûr, car, jusqu'à présent, les plans sociaux ne se sont jamais faits sans casse humaine, au moins pour les travailleurs les moins qualifiés, qui ont toujours peiné à retrouver un emploi et encore plus à ne pas subir une importante baisse de salaire. Monsieur le ministre, ma question est simple comment anticipez-vous le problème de la mutation nécessaire de l'emploi dans le cadre de la transition vers une industrie verte ? La parole

2 millions d'emplois industriels détruits depuis les années 1980, des usines qui ferment absolument partout, une part de la production industrielle dans la richesse nationale qui passe de 20 % à juste un peu plus de 10 %.

Les premières décisions que nous avons prises ont été de baisser l'impôt sur les sociétés, de diminuer les impôts de production, de mettre en place un prélèvement forfaitaire unique. Parce qu'il n'y a pas d'industrie sans capital, baisser la fiscalité sur le capital, c'est accroître l'industrialisation du pays. Voilà des vérités que personne ne voulait voir en face.

pour tous ceux qui travaillent dans les secteurs de l'hydrogène vert, des batteries électriques, des panneaux solaires, des véhicules électriques, pour favoriser la création d'emplois verts et industriels dans notre pays. Nous allons faire en sorte d'accélérer l'ouverture des usines et l'extension des usines vertes existantes pour accroître les relocalisations industrielles et les créations d'emplois. Quand ? Nous devons conjuguer croissance et et climat. Telle a toujours été la ligne de force du Gouvernement, de la Première ministre et du Président de la République. Les résultats sont là, nous allons accélérer.

un peuple refuse de se soumettre, il est vent debout contre une réforme dont il ne veut pas : le recul à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Face au mouvement social massif, qui porte l'exigence de retrait, face à une Assemblée nationale qui n'a voté la réforme ni en première lecture ni en commission mixte paritaire, vous vous enfermez, avec le Président de la République, dans un repli autoritaire, lourd de danger pour la démocratie. Vous avez affirmé vouloir aller au bout du cheminement démocratique. Quelle provocation ! C'est bien un chemin de croix auquel nous assistons, rythmé par les articles de la Constitution désormais connus de tous : 47-1, 44.3 et 49.3. Monsieur le ministre, comment parler de cheminement démocratique, alors que, depuis jeudi, le droit de manifester est mis en cause ? Le groupe CRCE demande que soit mis à l'étude le comportement des forces de sécurité depuis jeudi soir. Il ne s'agit pas de cautionner des dégradations, mais nous assistons à des violences policières et à des réquisitions inacceptables. Le maintien de l'ordre relève de votre responsabilité. Pour autant, l'ordre, ce n'est pas le matraquage et le gazage à tout va ! C'est savoir entendre la foule, l'opinion, le peuple qui dit non La colère est là, elle monte. La morgue et le mépris du chef de l'État ne passeront pas cette fois et la répression policière ne peut être la voie pour résoudre cette crise politique, sociale, très profonde. Le chef de l'État, droit dans ses bottes, ne veut ni dissolution, ni référendum, ni remaniement. Qu'il retire alors ce projet si injuste. Si, par malheur, M. Macron ne veut pas assumer cet échec, s'il s'y refuse, nous le contraindrons par la demande de référendum d'initiative partagée que nous avons lancée M. Macron, lors de son interview insipide et inutile, a affirmé choisir l'intérêt général. En réalité, entre le peuple et l'intérêt des riches, il choisit l'intérêt des riches. Demain sera une formidable journée, où un peuple uni, une foule immense, légitime, se lèvera pour défendre sa condition, pour défendre ses droits. Votre question ! Madame la Première ministre, il est encore temps : retirez votre projet !

Ce projet de loi faite suite à quatre mois de concertation. Il a donné lieu à plus de 175 heures de débat à l'Assemblée nationale et au Sénat et votre assemblée, le Sénat, l'a voté à deux reprises : une première fois en première lecture, après l'examen de chacun des articles, ... Par un vote bloqué ! ... une seconde fois, après que la commission mixte paritaire a abouti à une conclusion partagée.

rassurer les marchés financiers ! Il est nécessaire pour faire face aux déficits structurels et pour améliorer le système de retraite. Sa mise en oeuvre à la fin de l'année, lorsque le Conseil constitutionnel se sera prononcé, permettra de revaloriser les petites pensions, de mieux prendre en compte la pénibilité, mais aussi de mieux accompagner celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt.

madame la sénatrice, on soutient les forces de police placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Je profite de votre question pour saluer l'ensemble des forces de police et de gendarmerie, qui, par leur travail, par leur intervention, garantissent la sécurité et le maintien de l'ordre. C'est aussi l'expression de la démocratie et de la liberté.

Une exploitation et un surdéveloppement vampiriques, une exploitation non durable des ressources en eau, la pollution et le réchauffement climatique incontrôlé sont en train d'épuiser, goutte après goutte, cette source de vie pour l'humanité. » Ainsi s'exprime António Guterres dans l'avant-propos d'un rapport publié avant l'ouverture de la session inédite de l'ONU consacrée à l'eau, qui débute aujourd'hui. Les inondations au Pakistan en 2022 nous ont montré les conséquences du réchauffement de notre planète sur le cycle de l'eau : 33 millions de personnes concernées, 1 700 morts, 1,8 million d'hectares de terres agricoles dévastées. sur l'évolution du climat) montre que ces épisodes seront de plus en plus intenses et de plus en plus récurrents sous nos latitudes. Dans notre pays, l'hiver historiquement sec que nous venons de traverser nous montre qu'il est plus que jamais nécessaire de préserver cette ressource. C'est l'un des enjeux principaux de notre siècle. Ces impératifs nous pressent donc de modifier notre rapport à l'eau, nos modes de gestion afin d'en assurer la qualité, la quantité et le caractère renouvelable. Cette incertitude implique également de replacer l'eau au coeur de tous nos débats sur les changements climatiques. Le Gouvernement a annoncé dévoiler prochainement cinquante mesures relatives à la gestion de l'eau. Dans le cadre de cette journée de l'ONU consacrée à l'eau, madame la ministre, pouvez-vous nous en dire davantage sur le contenu de ces propositions visant à renforcer et à améliorer la gestion de l'eau dans notre pays afin d'en assurer la qualité et la quantité pour nos concitoyens ? La parole

de la cohésion des territoires, qui, comme vous le savez, est fortement investi sur ce sujet et qui rencontrera dans les prochains jours António Guterres pour fixer un agenda sur l'eau qui soit particulièrement ambitieux, tant internationale que nationale. Vous avez raison de mentionner également le rapport du Giec, qui confirme l'extrême urgence d'agir pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris en matière climatique.

a permis de doubler le rythme de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous continuerons d'agir. Je ne reviens pas sur le vote très large sur ces travées

État comme collectivités locales, mieux anticiper la diminution de la ressource en eau, mieux préparer les sécheresses à venir. C'est tout l'objet du plan Eau que la Première ministre et Christophe Béchu présenteront très prochainement, qui est une brique importante de l'ensemble de la planification écologique voulue par le Président de la République. Nous devons engager une réelle transition sur trois axes : la sobriété de nos usages- elle fera écho à la sobriété énergétique -, la garantie de l'accès à une eau potable de qualité

D'abord, il nous a dit que la majorité du pays, celle qui s'oppose à sa réforme, serait dans le déni de la réalité et dans l'ignorance- et que lui seul nous conduirait vers la lumière. C'est une insulte à l'intelligence des Français. Il nous a dit que les manifestants seraient noyautés par des factieux. Il est allé jusqu'à les comparer aux suprémacistes de Brasilia ou du Capitole. C'est encore une insulte. Il nous a dit que les syndicats auraient refusé de négocier. C'est un mensonge, a déjà répondu Laurent Berger.

Il nous a dit que les Français ne voudraient plus travailler et qu'il remettrait les bénéficiaires du RSA au travail. C'est une insulte. À la crise démocratique qu'il a approfondie, à la crise politique qu'il a ouverte, il a répondu par la perspective de nouveaux débauchages, sans doute parmi les députés qui n'ont pas voté la motion de censure. C'est une indécence. Il nous a dit vouloir taxer les entreprises qui rachètent leurs actions, sauver l'éducation, la santé et l'industrie, sans jamais préciser ni où, ni quand, ni comment.

La seule autocritique que vous nous concédez est celle d'une défaillance pédagogique. Vous voulez apaiser le pays ? Je le crois sincèrement. Mais il n'y a qu'une solution : rendez aux Français les deux ans de vie que vous leur volez

Je vous appelle « madame la ministre » parce que, en 2014, vous étiez ministre déléguée auprès de Marisol Touraine.

Sécheresse hivernale historique, inflation, difficultés de transmission des exploitations, élevages pastoraux en péril, prédation : la vulnérabilité du monde agricole est perceptible dans les discussions à bâtons rompus que nous avons avec les professionnels du secteur. Les réponses apportées par les autorités sont parfois insatisfaisantes et suscitent l'agacement, l'anxiété ou la résignation. À cela s'ajoute l'équation complexe sur les contours du futur dispositif d'affichage environnemental sur les produits alimentaires,

qui ont collecté des contributions jusqu'au 10 mars dernier, notamment sur les modalités d'affichage. L'analyse du cycle de vie est la méthode d'évaluation privilégiée pour classer les produits ou les services, en fonction des émissions de gaz à effet de serre, des atteintes à la biodiversité et de la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles que leur production a entraîné. En découle l'attribution d'une note, qui sera affichée sur les produits ou services, en rayonnage ou sur internet. Bien que ce dispositif réponde à une aspiration légitime des consommateurs, bon nombre de producteurs craignent qu'il ne soit inadapté à des produits locaux et artisanaux, à l'instar de ce qui avait été observé avec le Nutri-score.

L'information du consommateur sur les caractéristiques environnementales des produits est fondamentale pour faire évoluer nos modes de consommation. Nous voulons et nous devons permettre aux consommateurs de devenir des « consom'acteurs

Vous questionnez la méthode. Plusieurs expérimentations ont été conduites en 2021 sur les produits alimentaires et en 2022 sur le textile. Ma collègue Bérangère Couillard a réuni dès le mois d'octobre 2022 les associations de consommateurs, les ONG et les porteurs de ces expérimentations pour recueillir leurs attentes et leurs idées, afin de construire ensemble cet affichage environnemental. Priorité a été donnée aux produits alimentaires et aux textiles. L'objectif est, pour ces deux secteurs, qu'un affichage environnemental puisse être déployé dès le début de l'année 2024 par les entreprises volontaires, volontaires, avant de devenir obligatoire, comme le prévoit la loi. En ce qui concerne le secteur alimentaire, pas de découragement, pas de défaillance Ma collègue Bérangère Couillard réunira les parties prenantes le 27 mars prochain pour lancer une véritable concertation sur la première version du projet de méthode de calcul de l'affichage environnemental des produits alimentaires. La parole

Il faut le répéter : face aux mauvais procès qui sont faits à notre texte, le Sénat n'a pas bouleversé l'architecture du ZAN. Les cibles et les trajectoires sont intactes. Des ajustements, de la souplesse et des outils nouveaux étaient nécessaires pour répondre aux inquiétudes, voire à la colère, de certains élus locaux. Nous les avons écoutés et pris au sérieux. Longtemps muet sur le sujet, le Gouvernement dit aujourd'hui être prêt à adapter la loi. Il a longtemps sous-estimé, et sous-estime encore, le potentiel hautement inflammable du ZAN. Son approche comptable et recentralisatrice et l'absence d'accompagnement des collectivités face à ces nouvelles obligations inquiètent les élus de tous les départements et, ici, sur toutes les travées. Nos auditions nous ont convaincus qu'il était impératif d'apporter des réponses législatives à des questions aussi variées que celles qui portent sur le calendrier, les grands projets, la prise en compte des efforts passés, la garantie rurale, les communes littorales, les bâtiments agricoles ... Il fallait éteindre l'incendie.

lors de son discours de clôture du Congrès des maires de France, Mme la Première ministre a rappelé que le Gouvernement était prêt à un certain nombre d'évolutions, ... Prouvez-le ! ... comme la prise en compte des grands projets d'envergure nationale et la et la garantie rurale, à laquelle nous sommes tous attachés. Les propositions du Gouvernement ont été défendues par Christophe Béchu lors de l'examen de la proposition de loi sénatoriale sur le ZAN la semaine dernière. Vous le savez, monsieur le rapporteur, elles n'ont pas été retenues par le Sénat, qui a préféré ce que nous pensons être une trajectoire moins économe en termes d'artificialisation. Le Gouvernement considère aujourd'hui que le texte du Sénat ne permet pas de respecter la trajectoire ambitieuse de réduction de l'artificialisation que nous portons.

acceptable pour l'ensemble des acteurs- députés, sénateurs, associations d'élus locaux ou associations de défense de l'environnement

Ma question s'adresse au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La France est dans la rue pour manifester son désaccord profond avec le passage en force d'une réforme des retraites qu'elle rejette en bloc. Cette réforme n'est pas soutenable d'un point de vue humain et social, et son poids repose exclusivement sur les efforts des travailleuses et travailleurs.

qu'ils sont soumis à des conditions de plus en plus exigeantes et à des procédures toujours plus complexes, qui les maintiennent dans des situations de précarité et d'insécurité juridique et administrative inacceptables, une réforme de ces droits mérite d'être abordée avec sérénité et sérieux. C'est pourquoi, au vu du contexte actuel, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a demandé que ce projet de loi soit retiré de l'ordre du jour de notre assemblée. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les propos du Président de la République, qui semble annoncer une série de textes découpant votre projet de loi à la Quoi qu'il arrive, le Gouvernement peut et doit prendre rapidement les mesures qui s'imposent en matière de régularisation des travailleurs étrangers. Il n'est pas besoin d'une loi pour réviser au plus vite la liste des métiers en tension, dans le cadre d'une concertation avec les partenaires sociaux, ou pour donner des instructions aux préfets en faveur de l'admission au séjour des étrangers qui contribuent chaque jour à l'effort national- et cotisent pour nos retraites. Dans l'attente de mesures législatives permettant de sécuriser durablement leur séjour et leur emploi, il convient de ne pas maintenir ceux-ci dans une situation inadmissible de précarité et d'agir rapidement avec les outils existants. Monsieur le ministre, qu'attend donc le Gouvernement pour agir face à ces urgences ?

le 13 mars dernier, les 10 000 étudiants en sixième année de médecine étaient appelés à passer en centre d'examen des épreuves blanches en prévision du concours d'entrée à l'internat, prévu en juin prochain. Organisées par le Centre national de gestion, qui dépend de la tutelle de votre ministère, les épreuves ont vite tourné au fiasco : à répétition, impossibilité de valider les réponses, ralentissements, problèmes d'affichage, voire carrément déconnexion en cours d'épreuve. À tout juste trois mois des véritables épreuves classantes nationales, décisives pour le choix de la spécialité et du lieu d'exercice, ce coup d'essai constituait pourtant une occasion privilégiée pour les étudiants de se situer par rapport au niveau national et de tester les conditions qui les attendent. En outre, le concours répondait à de nouvelles règles d'organisation, suivant une méthodologie inédite. Les étudiants ne disposaient donc pas d'annales des examens précédents ni de supports pour s'entraîner. de gestion sont tout aussi lunaires. Plutôt que d'assumer la responsabilité d'un dysfonctionnement du système informatique, le centre préfère minimiser le problème et invoque une « incompréhension sémantique », suggérant que les épreuves auraient été non pas un véritable concours blanc, mais bien un simple test pour vérifier la performance du logiciel. On croit rêver ! L'Association nationale des étudiants en médecine de France demande que de nouvelles épreuves blanches soient organisées dans les meilleurs délais, sur une plateforme fiable et opérationnelle. À trois mois des épreuves de classement national, qui détermineront toute la carrière de nos futurs médecins, allez-vous enfin mener une politique ambitieuse d'investissement dans les moyens mis à disposition de nos étudiants ? Pouvez-vous garantir la totale fiabilité du support numérique des épreuves d'ici au mois

Lefèvre, pour la réplique. Nos étudiants en médecine ont connu beaucoup de déconvenues : des confinements à répétition, des enseignements à distance et du stress. Ils méritent davantage de considération. La France a un besoin urgent de nouveaux médecins, tout le monde le sait, particulièrement ici au Sénat. Nous devons donc tout faire pour mettre

Ce que les élus ne supportent plus, c'est de servir de défouloir. » Ces mots ont été prononcés par le président de l'association des maires du Morbihan lors de la présentation du nombre de démissions intervenues depuis trois ans. La situation est inédite dans le département : quatre élus municipaux démissionnent chaque semaine depuis 2020. Le mandat local n'attire plus. Le Morbihan n'est pas une exception : en Loire-Atlantique, un élu local démissionne chaque jour. Et nous savons que le phénomène est national. Plusieurs facteurs concourent à ces désengagements. Les élus subissent des violences de toute nature : physiques, verbales, les réseaux sociaux ... Et, trop souvent, les plaintes sont classées sans suite. Les élus sont résignés et exaspérés. L'empilement des normes et la lourdeur administrative découragent les bonnes volontés. Même les plus motivés ont du mal à concilier leur vie professionnelle avec

Au-delà de cette vague de démissions, la question se pose de la capacité même à maintenir un fonctionnement régulier des collectivités territoriales et à pourvoir aux fonctions d'élu. Madame la Première ministre, comment comptez-vous redonner des moyens et du sens au mandat de maire et, plus généralement, à celui d'élu local ? Ceux-ci sont les premiers remparts et les garants de notre démocratie.

Qui se réveille à cinq heures du matin quand la neige est tombée un peu trop fort pendant la nuit et que les routes sont encombrées ? Le maire ! Qui doit intervenir lorsque des conflits de voisinage peuvent dégénérer ? Le maire

En 2019, nous avons donc renforcé le régime de protection des élus, qui s'apparente désormais à la protection fonctionnelle applicable aux agents publics, notamment lorsqu'un élu fait l'objet de poursuites pour des fautes qui sont détachables de ses fonctions ou lorsqu'il est victime de violences ou d'outrages « à l'occasion ou du fait de ses fonctions Cette protection peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des élus qui seraient décédés dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine de ce décès.

cette situation contribuera à la crise profonde que connaissent nos institutions. Ne l'oublions pas, le maire est le représentant de l'État dans sa commune.

Depuis l'automne 2020, l'Arménie est en état de siège, après l'invasion de l'enclave arménienne de l'Artsakh par l'armée d'Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, qui s'en sert comme avant-garde pour poursuivre et achever l'éradication du peuple arménien entamée en 1915.

Les seuls qui aient droit de passage sont les Arméniens qui fuient la guerre, la famine et la misère, mais ils n'ont droit qu'à un aller simple, l'Azerbaïdjan comptant sur le départ des 120 000 Arméniens restants pour établir définitivement son joug sur ce territoire. là que d'une première étape pour rayer de la carte cette terre chrétienne qu'est l'Arménie, la plus ancienne du monde, aujourd'hui encerclée par l'expansion musulmane. Depuis nos villes des Hauts-de-Seine, qui accueillent une forte communauté d'origine arménienne, nous envoyons des vivres, des médicaments, et aussi des médecins, en partenariat avec l'association Lumière Française. Ainsi, nous essayons de forcer le blocus. Mais qu'attend le Gouvernement, au-delà des messages d'amitié, pour demander le respect des règles internationales et du droit des peuples ? L'Arménie, ce petit pays, porte les mêmes valeurs que les nôtres. nôtres. C'est vrai que l'Arménie, ce n'est pas l'Ukraine, et qu'on n'y trouve ni pétrole ni gaz, contrairement à l'Azerbaïdjan. L'Arménie n'a rien, hormis sa foi et son courage.

la France dénonce le blocage du corridor de Latchine par l'Azerbaïdjan et ses conséquences économiques et humanitaires. En effet, depuis cette date, la population ne peut plus circuler librement. Les vivres arrivent de façon parcimonieuse, grâce au Comité international de la Croix-Rouge, que la France aide, monsieur le sénateur, tout comme ses partenaires de l'Union européenne. Cette situation ne peut plus durer. La libre circulation doit être rétablie sans tarder et l'approvisionnement des populations du Haut-Karabagh doit être mieux assuré,

politique, qui est le seul possible. C'est un accord de paix que nous recherchons, et que l'Arménie recherche, monsieur le sénateur, avec son voisin. Je prévois de me rendre à Bakou et à Erevan dans le

Je le redis, monsieur le sénateur : nous sommes déterminés, je suis déterminée. La France agit, elle ne regarde pas ailleurs ; elle ne parle pas, mais elle

Dois-je rappeler que nous ne sommes à l'abri de rien ? Dans le pays le plus nucléarisé au monde, nous pouvons remercier tous les jours notre sûreté pour n'avoir connu, jusqu'ici, aucun accident nucléaire. L'IRSN est indépendant. Il exerce des fonctions d'expertise et de recherche, qu'il fournit à l'ASN. C'est l'ASN, en tant qu'autorité, qui prend les décisions. C'est basique, c'est efficace et c'est une nécessité absolue. Pourquoi casser ce qui fonctionne ? Pourquoi créer de la confusion, voire du désordre ? Les salariés de l'IRSN sont d'ailleurs sous le choc, KO debout. Sur quelle étude d'impact repose ce choix ? L'arrêt de quatre réacteurs à l'automne, à la suite de la détection de problèmes de corrosion sous contrainte,

reconnus internationalement. En matière de nucléaire, notre boussole doit être cette aiguë conscience des périls dont parle Edgar Morin. Votre volonté d'effacement de l'IRSN a

en matière énergétique, le Président de la République a un objectif ambitieux : faire de la France le premier grand pays à sortir des énergies fossiles et à reprendre en main son destin énergétique. C'est dans ce contexte que le Gouvernement travaille à un programme nucléaire de six nouveaux EPR 2 et à la mise à l'étude de huit réacteurs supplémentaires. C'est un projet pour notre indépendance énergétique ; c'est un projet pour la planète ; c'est un projet qui doit aussi nous permettre de reprendre le fil de la plus grande aventure industrielle française depuis les années 1970. Le conseil de politique nucléaire du 3 février dernier, qui s'est tenu sous l'égide du Président de la République et de la Première ministre, a mis à jour la feuille de route pour mobiliser tous les maillons de notre filière nucléaire. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a décidé le renforcement- le renforcement ! -de notre sûreté nucléaire en avançant sur le rapprochement de l'ASN et de l'IRSN. De quoi s'agit-il ? Très simplement, il est proposé d'élargir les missions de l'Autorité de sûreté nucléaire, en s'inspirant des modèles éprouvés des autorités de sûreté du Canada ou encore des États-Unis, en rapprochant la décision et le contrôle des missions d'expertise et de recherche. Il s'agit donc, au fond, de réunir sous la même bannière et sous le statut le plus indépendant qui soit, celui d'autorité administrative indépendante-

cette composition ASN-IRSN -deviendrait la deuxième autorité de sûreté du monde, au regard de ses moyens humains et financiers. Sa crédibilité scientifique serait en outre renforcée. Nous sommes donc bien loin des fantasmes et des modèles que vous évoquez.

ne délivreraient plus un seul laissez-passer consulaire et menacé de suspendre la délivrance des visas pour les Français souhaitant se rendre en Algérie. Je t'aime moi, non plus ! Où en sommes-nous, madame la ministre, de la main tendue et de cette repentance incessante envers l'Algérie ? Où sont les résultats ? La réforme de votre ministère, qui écarte des diplomates chevronnés, véritables négociateurs et bâtisseurs de ponts entre nos pays respectifs, commence à faire vaciller tout un édifice. À quand des mesures fortes pour une France forte et respectée ? Des mesures de rétorsion existent pourtant. Elles sont simples : suspendre la délivrance des visas aux Algériens souhaitant se rendre en France. Parallélisme des formes et égalité de traitement, ni plus ni moins

Comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien, sous l'autorité de Mme la Première ministre et de son homologue algérien, les 9 et 10 octobre 2022. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, le ministre de l'intérieur s'est ensuite rendu en Algérie le 17 décembre dernier. J'ajouterai enfin- vous l'avez oubliée -la visite en France du chef d'état-major de l'armée algérienne, une première depuis bien longtemps. Génial ! Monsieur le sénateur, il faut éviter de tomber dans le piège de ceux qui souhaitent faire échouer notre ambition. Ce n'est pas votre voeu, j'en suis sûre. Nous continuerons de travailler avec les autorités algériennes à la levée des difficultés constatées, car l'approfondissement de notre relation est dans l'intérêt de nos deux pays.

coopération soit cohérente, sur le retour en Algérie des Algériens en situation irrégulière, comme le droit le commande. Ce dossier fait partie de nos priorités immédiates. Nous y travaillons, notamment avec le président Tebboune, dont je suis sûre, monsieur le sénateur, que vous aurez noté avec intérêt les dernières déclarations. Enfin, je pense opportun de rappeler que la naïveté peut être considérée comme de la faiblesse. Non, madame la ministre, nous ne voulons pas d'une France qui se couche. Nous voulons une France qui se fasse respecter !

que lorsque le prix du baril baisse significativement, les prix à la pompe ne diminuent que très peu. Monsieur le ministre, il est d'usage de faire des comparaisons avec nos voisins européens. Aussi, je me suis permis d'observer la situation dans quelques pays

Comparaison n'est pas raison certes, mais comprenez que dans le contexte actuel de tensions économiques, sociales et maintenant politiques, nos concitoyens ont l'impression de ne pas payer le juste prix. Nos concitoyens, c'est évident, ne réclament pas un nouveau chèque carburant ; ce qu'ils veulent, c'est une véritable baisse des prix à la pompe. Monsieur le ministre, j'ai conscience que le prix des carburants est un mécanisme complexe. Il est temps cependant que les prix soient transparents et enfin cohérents avec les variations du prix du baril. Ma question est donc la suivante : que compte faire le Gouvernement, à très court terme, pour que les prix à la pompe reflètent enfin de manière plus visible les cours du marché du pétrole ? La parole

Le taux de change entre l'euro et le dollar peut également avoir un impact positif ou négatif sur le prix à la pompe. Je dois reconnaître que, ces derniers jours, les désorganisations dans les chaînes d'approvisionnement

à la pompe. Ce n'est pas normal. J'espère que le Gouvernement saura inciter à plus de transparence. Nous

La séance est reprise.

c'est avec plaisir que nous vous accueillons pour notre débat sur le rapport public annuel de la Cour des comptes, rendu public le 10 mars dernier.

Comme les années précédentes, un représentant de chaque groupe politique pourra s'exprimer au cours de ce débat. Notre choix d'un débat ouvert et pluraliste démontre l'intérêt que nous portons aux observations et aux recommandations formulées dans le rapport public annuel, qui rencontre chaque année un écho médiatique réel. choix traduit également notre attachement à la mission d'assistance du Parlement au contrôle du Gouvernement que notre Constitution confie à la Cour des comptes. Vos éclairages apportent un concours précieux à la mission de contrôle que nous avons tous ici à coeur de faire vivre et de renforcer. C'est vrai ! Cette année en particulier, monsieur le Premier président, au-delà de l'analyse de la situation d'ensemble des finances publiques,

Nous menons nos propres réflexions sur ce sujet- nous l'évoquions avant cette séance -dans le cadre notamment du groupe de travail transpartisan sur la décentralisation, qui a été mis en place le 5 octobre dernier.

de notre démocratie. Monsieur le Premier président, je vous invite maintenant à rejoindre la tribune

en application de l'article L. 143-6 du code des juridictions financières, j'ai eu l'honneur de vous remettre à l'instant, monsieur le président, le rapport public annuel de la Cour des comptes. Je vous remercie de l'accueil réservé à la Cour, qui traduit la qualité des liens qui unissent nos deux institutions. Vous savez à quel point, comme mes prédécesseurs, je suis attaché au rôle de la Cour des comptes à l'égard du Parlement. Depuis Philippe Séguin, qui a été Premier président jusqu'en 2010, la Cour des comptes se définit comme à équidistance entre le Gouvernement et le Parlement et sa mission d'assistance au Parlement est, pour nous, absolument essentielle. Je salue, d'ailleurs, l'attention du Sénat et l'organisation particulière de ce débat, qui permet à chaque groupe de s'exprimer. Ce n'est pas le cas dans l'autre assemblée et je pense que cette formule est extrêmement heureuse, en ce qu'elle permet un débat pluraliste sur nos travaux. J'ai grand plaisir à vous retrouver

du nom du ministre de l'intérieur de l'époque -fut, à l'évidence, une rupture historique avec la tradition centralisatrice française. Elle visait à donner aux collectivités territoriales la maîtrise de leur devenir et à leur permettre de rapprocher l'administration des administrés. Ce mouvement s'est concrétisé, dans un premier temps, par la fin de la tutelle des préfets sur les collectivités locales, par le transfert des fonctions exécutives vers les départements et vers les régions et par un nombre important

enjeux financiers, mais aussi institutionnels, et présenté une série d'exemples concrets montrant les forces et les faiblesses de cette organisation au regard de la qualité et de l'efficience des services rendus à la population.

Je me réjouis de cette évolution très positive et je remercie le Sénat de l'avoir particulièrement portée. Comme chaque année, le rapport public annuel est précédé d'un chapitre liminaire relatif aux finances publiques, dont la présence est à nos yeux absolument indispensable, tant la situation des finances publiques conditionne la conduite de la politique de la Nation- je ne sais pas comment on fait une bonne politique sans finances publiques saines -et tant son son actualité se révèle cruciale dans la période que nous traversons. On ne peut pas dire en effet que nos finances publiques soient dans le meilleur des états. Je commencerai donc par vous livrer nos grands messages sur la situation actuelle de nos finances publiques. Déjà dégradée avant la pandémie de covid-19,

La Cour préconise d'examiner sérieusement la qualité de la dépense publique pour réformer les politiques publiques et,, déterminer comment en maîtriser les coûts.

Le choc sur les prix de l'énergie et les conséquences de la guerre en Ukraine ont ramené la croissance à 2,6 %, en deçà des 6,8 % de 2021, une année, certes, de rattrapage exceptionnel par rapport à la terrible année 2020. L'économie française a heureusement montré des signes de résilience mais l'inflation s'est peu à peu imposée dans le paysage et devrait demeurer à des niveaux élevés en 2023, atteignant 4,2 % selon le projet de loi de finances initiale, soit un peu moins que la prévision qui fait consensus chez les économistes et que nous reprenons.

Hors crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), les mesures nouvelles en prélèvements obligatoires devraient rapporter au total 5,5 milliards d'euros en 2023, après une baisse de 5,7 milliards en 2022. baisses pérennes d'impôts ont été temporairement compensées par une hausse des recettes liées à l'énergie. Disons-le, c'est un dynamisme exceptionnel des recettes, notamment fiscales, qui a caractérisé les exercices 2021 et 2022, sans permettre pour autant une inflexion du déficit du fait d'un dynamisme tout aussi marqué des dépenses. cela ne vous surprendra pas -c'est pour nous le point le plus préoccupant, la dépense publique continue de croître à un rythme soutenu. Après avoir atteint 1 461 milliards d'euros en 2021, en valeur de 4,3 % en 2022 et augmenteront, selon les prévisions, de 3,2 % en 2023. À partir de 2020, le Gouvernement a mis en oeuvre ce qui a été appelé le « quoi qu'il en coûte », c'est-à-dire un ensemble de mesures importantes pour soutenir les ménages et les entreprises face aux effets de la crise sanitaire,

sortie, revendiquée, du « quoi qu'il en coûte », mais d'autres dépenses ont pris le relais, notamment pour atténuer la hausse des prix de l'énergie, pour un total de 25 milliards d'euros en 2022 et de 36 milliards en 2023. En parallèle, les dépenses publiques ont été mécaniquement alourdies par l'inflation.

énergétique brouille l'appréciation de l'évolution de la dépense publique totale. Même si l'on défalque ces mesures exceptionnelles, la dépense publique a continué de progresser en volume de 3,5 % en 2022 et de 0,7 % en 2023,

Là encore, les scénarios annoncés ne me paraissent pas satisfaisants. Les déficits ont atteint 6,5 % du PIB en 2021 et devraient se stabiliser autour de 5 % en 2022 et en 2023. C'est un ratio qui reste tout de même élevé, alors que la croissance va se tasser. Il en résulte une dette publique qui devrait atteindre 111 % du PIB en 2023, soit près de 14 points au-dessus de son niveau d'avant-crise. Cela représente 700 milliards d'euros supplémentaires. Prenons un peu un peu de recul historique. En 2000, c'est-à-dire lors de l'entrée dans l'euro- j'étais membre du Gouvernement, comme Alain Richard, ici présent -, la France et l'Allemagne avaient exactement le même taux de dette publique, soit 58,8 % du PIB.

-est, selon moi, tout à fait préoccupant et traduit une dégradation relative de nos finances publiques. Pour ma part, je n'ai jamais parlé de la France comme d'un pays en faillite. Je ne parle jamais de problème de soutenabilité de notre dette, car- fort heureusement ! -la France a une signature solide et reste arrimée à l'Allemagne. Toutefois, un pays endetté à l'excès ne dispose pas des marges de manoeuvre suffisantes pour investir à long terme dans son avenir, surtout si vous ajoutez à cela une hausse

c'est juste indispensable pour préparer l'avenir. Le panorama que je dresse est d'autant plus sérieux qu'un recul de la croissance est attendu en 2023.

J'insisterai sur un point : la situation et les perspectives des finances publiques appellent à assurer la soutenabilité de la dette publique ; c'est un enjeu de souveraineté. Voilà pourquoi nous plaidons pour un redressement de nos finances publiques sans tarder. Notre constat est simple et constant. Nous formulons trois objectifs pour la période 2023-2027. D'abord, réduire sensiblement les déficits pour repasser nettement et au plus tôt sous la barre des 3 car la plupart de nos partenaires européens n'attendront pas 2027 et feront le nécessaire dès 2025. Ensuite, amorcer sans tarder la décrue de la dette. Enfin, préserver notre potentiel de croissance. Quelles sont les pistes que nous proposons ? Nous en parlons souvent en commission des finances : il me semble que l'accent doit être résolument mis sur la maîtrise de la dépense. Cela passe par l'initiative d'une revue des dépenses, proposée par le ministre des finances, que j'approuve pleinement. Encore une fois, il s'agit non pas d'austérité, mais de regarder,

Autre point dont j'ai discuté souvent en commission des finances- je connais la difficulté politique du moment -, notre pays doit se doter rapidement d'une loi de programmation des finances publiques.

que la proposition de la Commission, qui met l'accent sur l'évaluation de la dépense publique ou encore l'appropriation nationale des règles de gestion des finances publiques, va dans la bonne direction.

Nous avons souhaité répondre à la question : le niveau de décentralisation et l'organisation territoriale française ont-ils permis d'atteindre les trois objectifs fondateurs des lois Defferre ? Ces objectifs étaient, je le rappelle, de renforcer la démocratie locale, rapprocher la décision politique et administrative du citoyen et d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la dépense publique. Notre rapport fait suite à un premier bilan de la Cour des comptes sur la décentralisation entre 2000 et 2010. Quelles conclusions tirons-nous ? Disons-le,

n'ont pas permis de remédier complètement aux défauts de notre organisation territoriale, faute d'une vision consensuelle entre les différents acteurs. En d'autres termes, l'ambition d'ouvrir un acte III ne s'est pas matérialisée par la reprise du processus de décentralisation de manière constante.

hésitant et même parfois contradictoire. J'en donnerai quelques exemples : la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite loi RCT, a rationalisé l'intercommunalité et a créé les métropoles,

loi 3DS repositionnent les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au service de leurs communes membres et développent la différenciation et l'expérimentation.

qu'un premier mouvement a cherché à renforcer l'échelon intercommunal et celui des régions, avec les grandes régions et qu'un second mouvement est au contraire revenu sur la demande de proximité, donc sur le rôle des communes et des départements.

pays comptait 34 955 communes pour une population moyenne d'environ 2 000 habitants, ce qui est bien inférieur à celle des communes de nos pays voisins. Vous le savez aussi bien que moi, dans le domaine de l'action publique, une taille critique est souvent nécessaire en matière de portage d'investissements lourds et structurants ou de prise en compte de la complexité juridique et financière de la gestion locale. La promotion des fusions de communes depuis la loi de 2015 a connu un succès très relatif. Le dernier point de notre diagnostic concerne l'État. Il nous semble que l'organisation de ses services n'a pas été adaptée pour tenir compte de l'évolution de la carte et des compétences des collectivités. Disons-le clairement, on a trop désarmé l'État déconcentré la baisse des effectifs a d'abord été le fait de l'échelon déconcentré, et non de l'administration centrale. Nous avons le sentiment-

clair, des compétences de plus en plus imbriquées et exercées par plusieurs niveaux de collectivités, d'où des mécanismes de coordination coûteux et rarement efficaces, un État très demandé, mais qui n'a pas la capacité de répondre

plusieurs coups de projecteurs sur des politiques qui illustrent ces aspects divers. Nous nous sommes ainsi intéressés au développement économique des territoires et à l'action sociale envers les publics les plus fragiles. On voit bien que l'on a des chefs de file, la région d'un côté, le département de l'autre, qui ne sont pas totalement reconnus comme tels, avec un enchevêtrement d'interventions et de compétences. C'est pourquoi nous appelons à renforcer cette dimension. Nous avons également pris acte d'aspects plus positifs, comme la décentralisation scolaire, qui a indéniablement permis d'améliorer les conditions matérielles d'accueil des élèves dans les collèges. un certain nombre de problèmes en matière de culture, de tourisme, de gestion quantitative de l'eau ; pour cette dernière, nous devrons renforcer le rôle de pilotage des communes. J'en viens à la gestion des déchets ménagers. La mise en La mise en place d'une économie circulaire impose d'associer davantage les filières de production, mais aussi les ménages à la prévention, au réemploi et au recyclage. Enfin, nous avons identifié des domaines de compétences un peu bizarres dans le sens où ils ne sont ni décentralisés ni clairement partagés et dans lesquels l'intervention des collectivités territoriales est à la fois de premier plan et confrontée à des défis croissants. Le premier d'entre eux est l'accès aux soins de premier recours. En la matière, les collectivités ont parfois pris, de manière spontanée

rapport invite à poser les bases d'une nouvelle étape de la décentralisation pour revoir la répartition des compétences entre l'État et les différents échelons de collectivités locales et pour doter chaque échelon des moyens lui permettant de les assumer dans les meilleurs objectifs d'efficacité. Il y a une réflexion à mener sur les institutions nous savons évidemment qu'il est tout sauf simple de réaliser la grande ambition d'un véritable acte III ou IV de la décentralisation. Néanmoins, et c'est notre message, on ne peut pas se satisfaire du. N'en restons pas là Nous proposons, pour le court et le moyen terme, plusieurs directions : simplifier le partage des compétences et responsabiliser les acteurs, ce qui est une priorité ; approfondir la coopération intercommunale et mieux l'articuler avec le rôle des communes ; renforcer la position de chef de file en matière de politiques partagées, surtout quand le nombre d'échelons est important ; préciser les modalités de coopération en évitant les concurrences inutiles ; utiliser effectivement la différenciation territoriale et les expérimentations pour tester des organisations plus efficaces et mieux adaptées à la diversité des situations locales. Nous réaffirmons en outre l'importance du rôle de l'État. Il doit plus que jamais assurer la fonction stratégique de régulateur et de partenaire des collectivités. collectivités. Le besoin d'État est très fort dans les territoires ; nous l'avons constaté à l'occasion de la crise sanitaire. L'État est attendu dans un rôle puissant de stratège des politiques nationales et de partenaire des collectivités. C'est pourquoi nous appelons à un réarmement de l'État déconcentré.

l'adaptation des politiques publiques au changement climatique. Le choix de présenter un rapport public annuel thématique est une manière non seulement de nous montrer davantage encore au rendez-vous des préoccupations de nos concitoyens et de leurs représentants, mais aussi de rendre des éclairages plus exhaustifs

qui sont, bien sûr, soumis à réfutation, comme tout élément du débat public. Il faudrait tout de même réapprendre, dans notre pays,

qui suscitera- j'en suis sûr -de nombreuses observations de la part de mes collègues. Avant d'aborder le thème de la décentralisation, je note que le rapport conserve une tradition : celle de consacrer sa première insertion à la situation de nos finances publiques. La Cour rappelle ainsi que la croissance s'est élevée à 2,6 % en 2022 et estime qu'elle devrait s'établir à seulement 0,5 % en 2023, soit en dessous de l'hypothèse gouvernementale de 1 %. Ces chiffres traduisent clairement le ralentissement de notre économie. Le déficit public atteindrait 5 % du PIB en 2023 et la dette publique 111,2 % du PIB. Les dépenses publiques ont, certes, progressé sous l'effet de l'inflation et des mesures de soutien à l'économie et aux ménages, ce qui explique en partie ces chiffres, mais, comme le note aussi la Cour, entre 2019 et 2023, les baisses discrétionnaires de prélèvements obligatoires ont représenté à elles seules un point de déficit public. Le projet de loi de programmation des finances publiques n'a toujours pas été adopté par le Parlement. La Cour note que celui-ci repose sur des hypothèses macroéconomiques très optimistes et estime, rejoignant ainsi la majorité sénatoriale, qu'il n'est pas suffisamment ambitieux en matière de baisse des dépenses. Je formule le voeu que la Cour tire aussi les enseignements de ses constats sur les prélèvements obligatoires pour observer que le projet de loi de programmation ne repose que sur une jambe, celle de la maîtrise des dépenses, sans jamais interroger le volet recettes. Nous aurons à en reparler dans les semaines et les mois à venir. à présent évoquer le bilan que dresse la Cour de la décentralisation. Le rapport montre que si les dépenses de fonctionnement et d'investissement des collectivités territoriales ont augmenté depuis le premier acte de la décentralisation, cette hausse s'explique par les transferts successifs de compétences et la recherche d'amélioration des services publics. La Cour reconnaît par exemple que la décentralisation a permis que la décentralisation a permis d'améliorer les conditions matérielles d'accueil des élèves dans les collèges- on pourrait aussi parler des écoles et des lycées -, même si les départements sont désormais confrontés aux enjeux de rénovation du bâti scolaire, notamment en matière d'efficacité énergétique : cette question est précisément l'objet d'une mission d'information du Sénat dont les travaux viennent d'être lancés.

regrettaient l'absence de réflexion sur la pertinence de l'action de l'État en faveur de la création dans les territoires, qui pourrait s'apparenter à un renouvellement automatique des aides habituellement versées, à l'image d'une dépense de guichet. De manière générale, qu'il s'agisse de l'appui au développement économique dans les territoires, de la gestion de l'eau ou des déchets ou encore des politiques sociales, sujet sur lequel nos collègues rapporteurs spéciaux de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » se sont largement penchés- la commission des affaires sociales a fait de même -, la Cour appelle à la clarification des compétences non seulement entre collectivités, mais aussi avec l'État. l'État. Globalement, le poids des dépenses locales dans le PIB demeure inférieur à la moyenne européenne. Comme le souligne la Cour, la France reste finalement un pays peu décentralisé. Pour en venir plus précisément aux finances locales, qui font l'objet d'un développement spécifique, le principal enjeu me semble résider moins dans le niveau des dépenses des collectivités que dans le mode de financement, ce dernier apparaissant de plus en plus inadapté. En effet, la substitution progressive aux ressources provenant de la fiscalité locale de parts d'impôts nationaux a distendu le lien qui existait entre les collectivités territoriales, pourvoyeuses de services à la population et aux entreprises, et ces derniers. Les dotations de l'État sont trop complexes et leur effet péréquateur est insuffisant. Le dispositif actuel manque de prévisibilité et de lisibilité pour les élus comme pour les citoyens. Les constats du rapport public rejoignent ceux de l'enquête de la Cour sur les scénarios de financement des collectivités territoriales demandée par la commission des finances en application du 2° de l'article 58 de la loi

sont partagés par l'ensemble des acteurs, élus locaux et parlementaires. La question qui doit désormais être posée est celle des mesures à mettre en oeuvre. Or nombre de sujets à trancher ne sont pas consensuels et mériteront dans les mois à venir d'être étudiés par le Sénat pour tracer des pistes concrètes : la frontière entre autonomie fiscale et financière et la place qui doit être faite à la première les modalités de compensation des transferts de compétences et des réformes de la fiscalité locale, la compensation au coût historique n'étant pas soutenable dans certains domaines et pour certains territoires le dynamisme des recettes qui doit être envisagé au regard de celui des charges. Aujourd'hui, le mode de financement des collectivités est trop souvent décorrélé de leurs charges et, plus fondamentalement, des missions qu'elles exercent et de la qualité des services publics. La question de l'éventuelle contribution des collectivités au redressement des finances publiques ne pourra être posée qu'une fois ces questions préalablement tranchées. Par ailleurs, il me semble indispensable d'avoir une approche différenciée de la situation financière des collectivités. La Cour souligne de manière régulière la bonne santé financière des collectivités, mais les écarts mais les écarts entre catégories de collectivités et au sein d'une même catégorie sont trop importants pour ne pas être pris en compte. En conclusion, En conclusion, le temps qui m'est imparti est trop court pour commenter l'ensemble des contributions particulièrement riches de ce rapport, qui se penche sur sept politiques sectorielles. Il n'est pas possible de porter une appréciation sur les nombreuses recommandations formulées par la Cour, qui dépassent largement l'analyse purement financière. La commission des finances, par ses rapporteurs spéciaux, qui suivent chacune des politiques publiques, tirera- soyez-en sûr, monsieur le Premier président -le meilleur profit de ces contributions, sur des sujets souvent abordés au moment de l'examen des projets de loi de finances. La parole

Merci comme chaque année, j'ai pris connaissance avec grand intérêt du rapport annuel que la Cour a publié le 10 mars dernier. Comme de coutume, ce rapport fait tout d'abord un point sur la situation

Elle pointe un risque de divergence entre plusieurs groupes de pays, la France appartenant à celui des pays les plus endettés et aux déficits les plus élevés. À partir de ce constat, elle appelle à un plus grand effort de maîtrise des dépenses publiques. Comme vous l'observez, monsieur le Premier président, la sphère sociale a déjà agi en la matière, au travers de la réforme de l'assurance chômage et, plus récemment, de la réforme des retraites. avoir des échanges, afin de déterminer si c'est toujours dans le domaine des finances sociales que vous distinguez des axes prioritaires de maîtrise de la dépense publique. En dehors de ce chapitre traditionnel, le rapport annuel prend la forme d'un bilan thématique consacré à la décentralisation, quarante ans après les lois Defferre. Il s'agit évidemment d'un sujet auquel le Sénat, représentant des collectivités territoriales, ne peut qu'être sensible. Je me suis tout particulièrement intéressée au chapitre relatif aux politiques sociales décentralisées. Les politiques de solidarité, dont le département est chef de file, représentent un volet important de la décentralisation, avec pour philosophie de mettre en oeuvre les dispositifs destinés aux publics vulnérables au plus près de leurs bénéficiaires. Les attributions des départements s'adressent principalement à quatre catégories de publics : l'enfance en danger ; les personnes en situation de pauvreté ou de précarité ; les personnes âgées dépendantes ; les personnes en situation de handicap. s'organisent notamment autour de prestations monétaires dont les caractéristiques principales sont définies à l'échelle nationale : le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Les départements doivent consacrer une part croissante de leurs dépenses de fonctionnement à ces allocations individuelles de solidarité, et leur reste à charge s'est creusé du fait de l'inadaptation des mécanismes de financement au dynamisme de ces dépenses. Dès l'origine, ces politiques ont souffert de la tension entre le caractère nécessairement national de la solidarité, corollaire du principe d'égalité, et la libre administration des collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences. Cette tension reste à ce jour irrésolue, ce qui a des conséquences sur l'efficacité des politiques et la qualité du service rendu aux usagers, et explique que la décentralisation n'ait pas tenu toutes ses promesses. La Cour met en évidence les enjeux de coordination qui résultent de la pluralité des intervenants : les départements, l'État, mais aussi le bloc communal, avec les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, la sécurité sociale, notamment ses branches famille et autonomie, et le service public de l'emploi. Ces acteurs interviennent indépendamment les uns des autres et le rôle de chef de file du département est, en réalité, peu opérant. La Cour des comptes formule ainsi des recommandations visant à rationaliser le déploiement des politiques sociales dans les départements, à en améliorer les outils de gestion et à en réformer le financement. En matière d'insertion et de lutte contre la pauvreté, le projet France Travail du Gouvernement vise à répondre à une partie des préoccupations de la Cour, en associant les régions et les départements autour du service public de l'emploi. Ce sera l'un des enjeux du projet de loi pour le plein emploi que le Gouvernement a annoncé pour l'été La commission des affaires sociales sera particulièrement attentive aux ambitions exprimées dans cette réforme en matière d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Ces dernières années, l'État a fait preuve d'une volonté de s'engager davantage dans l'animation de ces politiques, voire d'en recentraliser certains pans, à l'image de l'expérimentation du transfert à l'État, dans dans quelques départements volontaires- soumis, il est vrai, à de fortes contraintes financières -, du financement et de la gestion du RSA. Une démarche de contractualisation entre l'État et les départements a été mise en oeuvre dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte Par ailleurs, après avoir renoncé à son projet de revenu universel d'activité, le Gouvernement a récemment lancé plusieurs chantiers concomitants dont la cohérence ne se dégage pas encore avec clarté, le « RSA sous conditions » et le projet de « solidarité à la source », qui doivent donner lieu cette année à des expérimentations dans plusieurs territoires. J'indique que la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) conduira en parallèle une étude des conditions préalables à la mise en place de la solidarité à la source et de ses implications. Il apparaît donc que nous n'avons pas fini de tâtonner à la recherche de la bonne formule en matière de décentralisation des politiques de solidarité. En tout état de cause, il est indispensable que les collectivités intéressées soient associées à la conception de l'architecture de ces politiques. Je conclurai mon propos en remerciant la Cour des comptes de la qualité de ses travaux

Le constat de la situation extrêmement dégradée des finances publiques de notre pays est posé dans cet hémicycle depuis déjà plusieurs années. On ne peut que saluer la clarté de vos propos sur le sujet, monsieur le Premier président : « La France ne peut pas continuer sur cette voie, qui la distingue de ses partenaires européens. Il nous faut impérativement agir, faute de quoi tout cela pourrait se terminer très mal. En détail, que dites-vous ? Incontestablement, la situation de nos finances publiques est l'une des plus dégradées au sein de l'Union européenne. Alors que nous étions entrés dans la crise déjà affaiblis, le Gouvernement a fait le choix, à partir de 2020, de mettre en oeuvre diverses mesures pour soutenir les ménages et les entreprises face aux effets de la crise sanitaire, mesures prolongées par des dépenses de relance dès l'automne 2020.

Alors que l'année 2023 aurait dû être marquée par la fin du « quoi qu'il en coûte », nous continuons à mettre en oeuvre des mesures, insuffisamment ciblées, dont nous n'avons plus les moyens. Le résultat, c'est un déficit public qui, après avoir culminé à 6,5 % du PIB en 2021, devrait encore atteindre 5 % du PIB en 2023

Nous divergeons incontestablement de la courbe de nos partenaires, et cela nous affaiblit. Un désendettement maîtrisé est impératif pour assurer la soutenabilité de notre dette publique. Certes, son taux est encore arrimé à celui de l'Allemagne, mais pour combien de temps ? C'est le premier enjeu de souveraineté ! Hors dépenses exceptionnelles, la hausse de nos dépenses atteint 3,5 % en 2022 ; elle sera encore de 0,7 % en 2023. Rappelons que l'objectif était de 0,6 % par an jusqu'en 2027 : on en est donc loin Le budget pour 2024 devra donc être plus exigeant sur ce front que celui de 2023. À 58 % du PIB, la France a le taux de dépenses publiques le plus élevé de la zone euro. Pour autant- c'est à la fois un paradoxe, une incompréhension et une difficulté démocratique -, cela ne s'accompagne pas d'un haut niveau ressenti de performance des services publics. En outre, un pays endetté à l'excès ne peut pas financer la préparation de son avenir. Notons que l'endettement des collectivités territoriales est, quant à lui, très faible- moins de 9 % de l'ensemble -, confirmant que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faudra accomplir l'essentiel des efforts. Il faudra des milliards pour la transition environnementale et énergétique, pour combler notre retard en matière d'innovation et de recherche, pour renforcer notre politique industrielle ou encore notre système hospitalier. Tout cela, le pays en a besoin. Mais aujourd'hui, il ne s'en donne pas les moyens. La fuite en avant n'est plus possible

ce qui signifie que ses prévisions sont fragiles et que le moindre accroc remettrait en cause le passage sous la barre des 3 % à la fin du quinquennat. Mais il est également peu ambitieux de vouloir revenir tout juste sous 3 % en 2027, alors que la quasi-totalité des pays de la zone euro devraient repasser sous cette barre dès 2025. Nous sommes en train de décrocher sur le front du déficit et de la dette, et cela va finir par se voir. Il y a trois leviers pour réduire les déficits, comme vous le rappelez utilement dans votre rapport, monsieur le Premier président. Le premier consiste à espérer que cette réduction provienne essentiellement de la croissance. Renforcer celle-ci y contribue évidemment, et c'est pour cela qu'il nous faut investir. Mais nous entrons dans une période de croissance modérée, et ce levier ne sera pas suffisant. Le deuxième consiste à augmenter les impôts. C'est particulièrement compliqué dans un pays où les prélèvements obligatoires sont déjà très élevés- 45 % -et où le consentement à l'impôt est faible. La troisième voie consiste à maîtriser intelligemment les dépenses. Il faut commencer par là. Il faut insister sur la qualité de la dépense publique. C'est le chemin dans lequel nous voulons nous engager.

Avec un poids relatif de la dépense publique locale très modéré- 19 % de l'ensemble, alors que la moyenne européenne se situe à 34 % -, nous restons un pays marqué par notre tradition centralisatrice. La décentralisation est un mouvement historique qui doit être non pas remis en cause, mais remis sur pied, consolidé. On peut surtout parler d'un essoufflement de la décentralisation et de contradictions qui ne sont pas propices à la meilleure efficacité de l'action publique, comme vous le soulignez dans votre rapport. Plusieurs réformes de l'organisation territoriale ont été menées depuis 2010, sans rien clarifier, sans marquer une vraie décentralisation politique aboutie. Les faiblesses de la décentralisation sont en partie dues au brouillage des compétences entre État et collectivités. Il faut lancer un nouvel acte de la décentralisation qui clarifie la répartition des compétences, avec une véritable liberté locale quant à leur exercice, et veille à doter chaque échelon des moyens requis pour assumer Le Sénat s'y emploie, sur l'initiative du président Larcher, qui a mis en place un groupe de travail dont les propositions seront rendues d'ici à la fin du printemps. Oui, il convient de redéfinir le mode de financement des collectivités territoriales comme vous le préconisez. Vous avez présenté à cette fin des orientations devant notre commission des finances.

et assure le lien de proximité, tellement indispensable, que beaucoup s'emploient à distendre, voire à rompre depuis bien des années. Dès lors, non à la réduction autoritaire du nombre de communes, qui remplissent une mission essentielle pour un coût modique. Au contraire, il faut les renforcer. Ce n'est pas seulement affectif ; c'est efficace

notre fiscalité : réduire significativement la dépense fiscale et sociale ; engager une revue des dépenses publiques permettant de limiter la dépense inefficace ou injustifiée débureaucratiser et différencier les approches, et limiter la place de l'administration administrante ; s'engager à mettre en place une règle d'or, dans le cadre d'une nouvelle gouvernance européenne ; décentraliser vraiment. en donnant pouvoir, moyens et liberté locale aux collectivités ; en recentrant l'État sur ses seules dépenses régaliennes ; en imposant des blocs de compétences exclusives et une autonomie fiscale pour chaque échelon de collectivités ; en engageant une véritable politique d'aménagement du territoire qui s'attaque à la rénovation de nos infrastructures et, plus largement, confronte les enjeux de l'eau et de la mobilité.

le rapport de la Cour des comptes agit chaque année comme une piqûre de rappel : il nous renvoie à la situation très dégradée de nos finances publiques. Ce n'est pas seulement la photographie à la date d'aujourd'hui qui doit nous alerter ; c'est aussi le film de la dernière décennie. La photographie, d'abord, c'est un déficit à 5 % du PIB et une dette de 3 000 milliards d'euros : la situation demeure très préoccupante. Certes, le Gouvernement était parvenu à sortir le pays de la procédure pour déficit excessif avant la crise sanitaire. Mais le retour dans les clous de Maastricht, conformément à nos engagements européens, n'est pas envisagé avant 2027. Le film de la dernière décennie, ensuite. Depuis 2010, la dette publique de la France est passée de 85 à plus de 110 % aujourd'hui, alors que l'Allemagne, qui en était au même point que nous, a su ramener sa dette à 70 % de son PIB dans le même intervalle. Le décrochage d'avec nos voisins allemands se creuse et nuit à notre crédibilité sur la scène européenne. Au fond, il n'y a qu'une explication valable pour ce décrochage. La dépense publique n'a jamais cessé de croître, et elle a toujours crû plus vite que les recettes. Je ne fais pas ici allusion à la période de crise sanitaire. Le « quoi qu'il en coûte » était nécessaire pour préserver nos entreprises et nos emplois. Mais cette parenthèse est close, et nous devons désormais remettre de l'ordre dans nos comptes. C'est pourquoi je salue la décision du Gouvernement d'engager une vaste revue des politiques publiques, afin d'identifier les économies possibles dans chaque domaine de l'action publique. Cette analyse est nécessaire pour que nous tenions l'objectif d'un déficit à 3 % du PIB en 2027. Il est bien logique que les collectivités territoriales soient intégrées à cette vaste revue globale. Il en faudrait plus pour effrayer les élus locaux, eux qui sont tenus de présenter, chaque année, des comptes à l'équilibre. Cependant, il me paraît important de rappeler quelques vérités, afin de ne pas se tromper de problème.

Elles représentaient 8 % du PIB en 1980, contre 11 % aujourd'hui. Toutefois, cette augmentation apparaît bien limitée si on la met en regard de toutes les compétences qui ont été transférées de l'État aux collectivités. Ensuite, il y est rappelé que la France reste un pays très centralisé. Globalement, la part des dépenses locales dans le PIB demeure en France inférieure à la moyenne européenne, qui se situe à 18 % du PIB.

Il faut se rendre à l'évidence : nous ne rétablirons pas les finances publiques en contraignant davantage les collectivités locales. De même, ce n'est pas en recentralisant certaines compétences que nous améliorerons la qualité des services publics.

Il faut rapprocher l'endroit où la décision est prise de celui où elle est appliquée. Il faut rapprocher le décisionnaire du bénéficiaire pour améliorer la qualité des services publics. Je l'ai dit : le rapport annuel de la Cour des comptes est éclairant à bien des égards. Mais la préservation des libertés locales ne doit pas être tranchée selon le seul angle budgétaire. Bien souvent, la respiration démocratique échappe aux chiffres. C'est pourquoi nous considérons qu'il faut poursuivre la trajectoire de décentralisation, à la fois pour dynamiser les territoires et pour réduire les dépenses publiques. La parole

Monsieur le Premier président de la Cour des comptes, je vous écoute et vous lis avec attention et intérêt. La décentralisation est sans doute l'un des outils qui renforcent nos capacités à agir. Encore faut-il réellement la promouvoir et non pas, sans cesse, notamment du côté de Bercy, vouloir contrôler l'action territoriale et la contraindre financièrement. La crise démocratique n'est pas uniquement due à l'actuelle réforme des retraites. Elle est le fruit d'une absence de vision partagée au sein de notre société du pays que nous voulons construire, ainsi que d'un manque de collaboration avec les corps sociaux et les élus locaux. Les résultats de notre pays sont contrastés, comme vous l'indiquez, et ce n'est pas vrai seulement d'un point de vue financier. Le contraste est aussi démocratique et social, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est perçu comme juste et ce qui ne l'est pas. Les Françaises et les Français subissent les inégalités brutales de notre société. Ils savent que les entreprises du CAC 40 reversent des dividendes records à leurs actionnaires sans pour autant rectifier les écarts de rémunérations, que ce soit entre les femmes et les hommes ou entre les bas et les hauts salaires. Ils voient des services publics en difficulté. Le regard qu'ils portent sur notre société est marqué d'un sentiment d'injustice, l'attente vis-à-vis des collectivités croît à mesure que la confiance envers l'État décroît. La Cour des comptes a choisi de travailler, pour son rapport annuel, sur le bilan de la décentralisation. C'est un sujet qui nous anime et nous passionne. Pour ma part, je veux affirmer une certitude, qui se traduit d'ailleurs dans votre rapport, monsieur le Premier la décentralisation est un de nos meilleurs atouts face aux crises. Elle a permis d'immenses progrès dans de nombreux domaines, en rapprochant des citoyens la gestion et la décision. En effet, la démocratie s'enrichit du contrôle direct et de la proximité. À la manière d'un Georges Perec, je voudrais un instant vous dire : « Je me souviens. Je me souviens que, dans les années 1970, pour le jeune banlieusard que j'étais, le cinéma, la musique, les spectacles n'étaient qu'à Paris, alors qu'aujourd'hui les festivals couvrent tous les territoires et participent au dynamisme de nos régions. Je me souviens du 6 février 1973, date de l'incendie dramatique du collège Édouard-Pailleron, à Paris. La confiance envers l'État avait brûlé aussi vite que ce bâtiment, alors qu'aujourd'hui les départements, véritables acteurs de la communauté éducative, consacrent aux collèges en moyenne 6 % de leur budget, le double de ce qu'ils investissaient au début des années 1980.

mais l'État jacobin et ses services centraux ont-ils, au fond, jamais renoncé à faire rentrer dans le rang la capacité d'initiative des élus territoriaux, que les lois de décentralisation avaient stimulée et que la Constitution a reconnue ? Je me souviens que François Mitterrand disait à raison : « La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. »

et l'État stratège ! Je me souviens enfin du cycle de l'eau, que l'on m'expliquait à l'école. Aujourd'hui, le dérèglement climatique a tout changé. La ressource abondante, dont on ne se souciait guère, est devenue un sujet majeur de préoccupation. Vous avez raison, monsieur le Premier président, de rappeler que l'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Alors que notre pays ne respecte pas ses propres principes sur le bon état de la ressource, il est aujourd'hui confronté à une réalité terrible : l'insuffisance quantitative, à laquelle nous ne sommes pas assez préparés. Les conflits d'usage se développent et les contradictions existent au sein même du Gouvernement : les priorités des ministres de l'environnement, de l'agriculture, de la santé ou encore de l'énergie divergent et ne semblent guère arbitrées. Ces conflits témoignent de la nécessité de nouvelles modalités de gouvernance démocratique,

encore et encore ceci : il est urgent d'agir ! Monsieur le Premier président de la Cour des comptes, la dette climatique coûte et coûtera plus cher que la dette financière. Surtout, elle ne se rembourse pas. Nous attendons avec impatience votre rapport sur le sujet l'année prochaine.

ans après le début du mouvement décentralisateur amorcé par la promulgation des lois Defferre, la Cour fait état d'un « élan à retrouver ce n'est pas là une surprise, mais un constat que nous faisons avec vous, car nous croyons qu'une vraie décentralisation est nécessaire et que l'engagement des élus locaux doit être au coeur de l'action publique.

La République, c'est la solidarité nationale. Et il ne faudrait pas que la décentralisation devienne l'alibi de son affaiblissement. » Monsieur le Premier président, le bilan que vous dressez de ces quarante au constat d'une absence de cap clair et lisible et d'un éparpillement des compétences, avec parfois un risque de chevauchement entre les différents niveaux de collectivités. Ce constat est resté le même depuis le rapport de 2009, car l'organisation des services déconcentrés de l'État a failli à s'ajuster aux évolutions- parfois erratiques, il faut le reconnaître -de la carte et des compétences des collectivités. L'architecture de financement est le reflet de cet éparpillement organisationnel. La Cour nous l'a montré à la fin de l'année dernière, à l'occasion d'un rapport qui mettait en lumière un système de financement à bout de souffle, souffrant d'un manque de lisibilité et de prévisibilité.

qui épouse cette nouvelle architecture. De ce point de vue, la position de l'exécutif est claire et va dans le bon sens. Elle s'articule autour des quatre principes suivants transférer des compétences ; accorder des ressources dynamiques et adaptées ; donner des capacités de différenciation, et j'insiste sur ce terme ; assumer les responsabilités qui vont avec.

un appel à la coconstruction, avec l'État, d'une décentralisation mieux adaptée à la réalité de ces territoires, une décentralisation qui conjugue la pleine égalité des droits avec la reconnaissance des spécificités et qui refonde la relation entre les territoires d'outre-mer et la République par la définition d'un nouveau cadre. Les signataires ont été reçus le 7 septembre 2022 par le Président de la République. Des travaux se déroulent actuellement au sein de chaque territoire autour de cette question, et un comité interministériel de l'outre-mer devrait se tenir à la fin de ce semestre, afin d'avaliser une première série de décisions. Monsieur le Premier président, je compte sur votre expertise, qui sera- j'en suis sûr -sollicitée pour que les collectivités d'outre-mer bénéficient d'une

dans leurs multiples et vaines tentatives de convaincre l'opinion de la nécessité de la réforme des retraites, le Gouvernement et ses alliés de la majorité sénatoriale ont souvent fait valoir la question de la dette. C'est précisément ce chantage qui a amené le Gouvernement à reprendre la rhétorique de François Fillon en 2007 sur le

Mais nous voyons clair dans le jeu du Gouvernement. Étant établi que les entreprises disposent toujours du levier du chantage à l'emploi et que le mouvement social est ignoré par ce gouvernement, il est aisé de deviner où l'exécutif compte réaliser l'essentiel de ces économies. je ne pense pas que les 160 milliards d'euros d'aides aux entreprises feront l'objet d'une refonte massive, afin d'éviter à nos concitoyens une cure austéritaire ... Reste désormais à savoir sur quoi repose cette nouvelle alerte sur la dette publique. Dans son rapport, la Cour des comptes critique le scénario d'évolution de la dette publique construit par le Gouvernement. Néanmoins, monsieur le Premier président, il comporte un impensé de taille.

Comme vous le savez, il existe une dynamique fondamentale entre la dette et l'inflation. Aussi, je m'étonne que cette question soit absente des discussions entre Bercy et la rue Cambon. L'inflation étant avant tout un phénomène redistributif,

et inférieur au taux d'inflation, alors le créancier ne peut pas compenser cette perte de valeur. Celui-ci ne peut alors qu'ajuster le taux des nouvelles émissions, ce qui ne règle pas le problème de la dette passée. Ainsi, l'inflation conduit souvent à une redistribution entre créanciers et débiteurs au profit des seconds. cela se vérifie particulièrement pour ce qui concerne la dette publique. Celle-ci est contractée très largement à taux fixe, et elle est « roulée ». De fait, le capital est remboursé par une nouvelle dette. Mais comme le capital remboursé est déprécié par l'inflation,

si la tension qui s'exerce sur les finances publiques ne peut pas être ignorée, il apparaît primordial d'explorer toutes les pistes d'assainissement, afin que celui-ci ne s'effectue pas au prix d'une nouvelle casse sociale que notre pays et nos concitoyens ne pourraient pas supporter.

mettre fin à un régime centralisé », « modifier profondément la répartition des pouvoirs entre l'État et les collectivités locales », donner à celles-ci la « maîtrise de leur devenir » et permettre de « rapprocher l'administration des administrés ». Belle promesse ! D'ailleurs,

Deuxième paradoxe : la décentralisation de certaines compétences s'est immédiatement accompagnée d'une recentralisation des ressources, avec à la clé des transferts de compétences sans moyens budgétaires propres.

Entre 2012 et 2022, nous avons assisté à une hémorragie des services déconcentrés de l'État, avec une coupe de 14 % des effectifs, soit 11 763 équivalents temps plein, des préfectures et des directions départementales et régionales. régionales. Mes chers collègues, quand l'administration territoriale de l'État disparaît, ce sont la cohérence, l'égalité et l'unité de la Nation et des services publics qui disparaissent avec elle.

! En opposant les échelons territoriaux faute de définition des coopérations intrinsèques aux enjeux du siècle et aux disparités territoriales, nos concitoyennes et nos concitoyens se sentiront démunis et dépossédés de leur capacité d'action et de leurs revendications légitimes.

56 % des masses d'eau de surface et 33 % des masses d'eau souterraine ne sont pas en bon état au sens de la directive communautaire sur l'eau. Pourtant, tous les échelons des collectivités sont mobilisés, dans une confusion déplorable.

Ces échecs créent des tensions sociales importantes. Des conflits d'usage émergent, la puissance publique n'étant pas aux rendez-vous. Il nous faut tirer les leçons du passé, consacrer le retour de l'État dans les territoires et- je vous le dis avec solennité -relégitimer la démocratie de terrain,

ans après la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, nous sommes invités à commenter la publication du rapport annuel de la Cour des comptes, qui dresse le bilan de la performance de l'organisation territoriale de la France. offre l'occasion de mesurer la qualité et l'efficience des services rendus à la population dans les domaines d'action publique partagés entre l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, mais également les organismes de sécurité sociale.

et les injonctions de la Commission européenne sur le choix des orientations stratégiques et budgétaires. Pour ma part, j'estime que l'équilibre des comptes est une nécessité, comme le soulignait Pierre Mendès France bien avant la signature du traité de Maastricht. Pour atteindre cet objectif, la réduction des dépenses n'est pas l'unique solution : on peut aussi jouer sur les recettes. Permettez-moi d'évoquer le fameux couperet de 3 % du PIB, limite vertueuse fixée comme objectif aux États membres de l'Union européenne. Comment ce chiffre a-t-il été choisi ? Une part de mystère demeure, mais il semble correspondre au niveau de l'érosion monétaire au moment de la signature du traité

seule une véritable nouvelle étape de la décentralisation permettra de remettre en ordre nos comptes publics. Si nous avons décentralisé, il y a toujours autant de ministères

Madame la présidente, monsieur le Premier président, mes chers collègues, depuis plusieurs années, la dette publique française file, malgré les mises en garde de diverses institutions nationales ou européennes. Si la crise du covid-19 a coûté cher, elle n'explique pas toutes nos difficultés. Les chiffres du commerce extérieur sont très inquiétants. Les taux d'intérêt remontent lentement, mais avec régularité. Le conflit en Ukraine pourrait durer encore plusieurs mois, voire plusieurs années, continuant ainsi de dégrader nos économies. L'inflation alimentaire et énergétique tire les prix à la hausse et pénalise les entreprises, les services publics et les consommateurs. De plus, il nous faudra suivre de très près, dans les semaines à venir, les conséquences sur les marchés de la fermeture

Comme le souligne la Cour des comptes, la situation des finances publiques restera en 2023 « parmi les plus dégradées de la zone euro, alors que la Commission européenne juge que les risques sont élevés sur la soutenabilité de la dette française à moyen terme En positivant, nous pourrions nous convaincre que la dette a servi à préserver notre modèle social, nos services publics et notre économie. Mais qu'en est-il réellement ? ? La crise sanitaire a révélé au grand jour l'état réel de l'hôpital public et les difficultés des soignants. Elle a montré les effets délétères de la mondialisation, notamment des pertes de souveraineté. La guerre en Ukraine a fait apparaître les limites de notre modèle d'armée. La crise énergétique a mis en lumière les renoncements de l'État en matière de nucléaire. Le changement climatique appelle des investissements massifs.

programmation militaire, nous mesurons les limites du modèle expéditionnaire et échantillonnaire français dans la perspective de la survenue de conflits de haute intensité : lacunes capacitaires, problèmes de stocks et de masse, extension de la guerre multichamps-multidomaines, concurrence industrielle étrangère de plus en plus rude Nos grandes compétences sont encore en France, notamment s'agissant de la dissuasion ; il nous faut impérativement les y maintenir. De même, préservons nos pépites technologiques des prédations étrangères, et soutenons-les dans leur croissance. Il y va de notre sécurité et de notre souveraineté,

Fractures territoriales, fractures sociales ... Quarante ans après les premières lois de décentralisation, dont la Cour dresse le bilan, les territoires sont, à juste titre, inquiets pour leur avenir. Comme de nombreux collègues, je le constate dans mon département. Je crois sincèrement que les Français demeurent très attachés à leur commune et à leur maire, échelons de proximité, qu'ils connaissent le mieux et dont ils ont pu apprécier le rôle durant la crise sanitaire. Pour autant, la succession rapide des dernières réformes a contribué à brouiller le paysage institutionnel local et les compétences de chacun. La dématérialisation a altéré le lien humain entre administration et administrés, tandis que l'État a progressivement réduit ses effectifs déconcentrés. Chez les élus, la fatigue législative et réglementaire est réelle. La voie de la réforme permanente et de l'inflation des normes, qui leur

Sinon, nous n'aurons plus de candidats pour faire vivre la démocratie locale. Qu'il s'agisse de la maîtrise des dépenses, de la préservation de notre souveraineté ou de l'avenir de la décentralisation, nous avons besoin d'un véritable État stratège avec une vision à long terme.

l'examen du rapport annuel de la Cour des comptes est toujours un moment important pour les parlementaires. Cette année, la Cour aborde un sujet auquel les sénateurs, représentants des territoires, prêtent une attention toute particulière : la décentralisation.

les compétences s'entremêlent toujours plus, les modalités de financement se sont complexifiées et, plus encore, l'État n'est pas au rendez-vous. Nous le constatons tous, dans nos départements : l'organisation de l'État reste en décalage avec le maillage territorial. Ainsi, la baisse très importante des effectifs des services déconcentrés de l'État s'est traduite par un désengagement de celui-ci dans les territoires,

Déconcentration et décentralisation doivent impérativement être coordonnées pour répondre à l'exigence de proximité de nos concitoyens. Nous voyons bien à quel point cette proximité est essentielle. les crises récentes ont mis en lumière, si besoin en était, le rôle essentiel des services publics et la nécessité de les renforcer en tout point du territoire. C'était bien là l'un des objectifs de la décentralisation telle que la voulait le président Mitterrand. L'acte I a d'ailleurs pleinement joué son rôle en renforçant la démocratie locale, en rapprochant la décision politique du citoyen et en donnant aux collectivités territoriales les moyens financiers et humains d'exercer les compétences transférées. Toutefois, après plusieurs réformes décentralisatrices, le message s'est brouillé. Si une clarification s'impose quant à l'exercice des compétences et la complémentarité des différentes collectivités- car nous savons bien que certaines compétences partagées donnent de meilleurs résultats -, la question des moyens des collectivités se pose avec une acuité particulière.

La Cour qualifie d'« inadaptée » la substitution progressive des ressources fiscales des collectivités par des dotations de l'État, tant la cohérence entre les recettes locales et les compétences exercées s'en trouve réduite. Les suppressions de la taxe professionnelle en 2011, de la taxe d'habitation en 2020 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2023, puis en 2024 illustrent parfaitement ce constat. Ces différentes réformes sont autant d'atteintes à l'autonomie financière et fiscale des collectivités. Elles ont en outre distendu le lien qui existait entre les communes et leurs administrés, utilisateurs des services publics locaux. Par ailleurs, le manque de lisibilité et de prévisibilité des finances locales, ainsi que la réduction des marges de manoeuvre des communes sont un frein important pour l'investissement public. communes y prennent pourtant- nous le savons bien -une très large part, en apportant un soutien indispensable à l'économie locale et à l'emploi. L'enchaînement des crises économique, sociale et sanitaire, ainsi que la forte inflation rendent nécessaire la refonte du financement de nos collectivités, afin de préserver le maillage territorial assuré par nos communes. Si j'ai un point de désaccord majeur avec la Cour, c'est bien au sujet de nos communes, qui sont l'échelon de proximité indispensable au maintien de la démocratie locale et doivent être préservées. En revanche, pour mieux fonctionner- le constat est clair -, l'organisation territoriale de notre pays requiert une articulation plus fine entre l'État et les collectivités.

Pas plus que les départements et les régions, les communes n'ont vocation à être les variables d'ajustement des comptes publics. Il nous faut donc renouer avec les objectifs initiaux de la décentralisation et instaurer un véritable dialogue de confiance entre l'État et les collectivités, dans le respect de la libre administration de ces dernières. La parole

Madame la présidente, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, avec ce rapport, la Cour nous alerte une fois de plus sur la situation dégradée de nos finances publiques et, plus significativement encore, sur la position tristement singulière de la France. Processus lent, longtemps imperceptible, notre déclassement s'accélère tout à coup sous le poids des contraintes extérieures et des incuries intérieures. Faute de temps, je n'évoquerai qu'un seul sujet, celui des finances des collectivités locales. Si je partage les constats de la Cour des comptes, je suis plus réservé sur ses préconisations. Dans sa rétrospective, celle-ci revient sur le remplacement de pans entiers de la fiscalité locale par des impôts nationaux, ce qui a eu pour effet de desserrer le lien entre taxation et représentation. Comme la Cour, je regrette que l'on ait cassé un ressort essentiel de la démocratie décentralisée : le consentement local à l'impôt. On a trop vite oublié que c'est à l'aggravation des déficits et de la dette publique et, plus généralement, à ce qui a été qualifié à peu près à peu près partout en Occident de crise de l'État-providence que l'on doit la poussée décentralisatrice du début des années 1980. Cette revanche du local

le flot croissant des exonérations et des dégrèvements et, plus généralement, le remplacement de la fiscalité locale par les mécanismes centralisés que sont les dotations budgétaires en ont décidé autrement. Loin de freiner la décrépitude du système fiscal local, l'introduction dans la Constitution d'un article consacré à l'autonomie financière des collectivités en 2003 n'a fait que réduire la libre administration à une simple liberté de gestion. La réforme de la fiscalité locale voulue, après bien d'autres, par Emmanuel Macron aurait pu combler un tant soit peu cette faiblesse. Or il n'en est rien. C'est pire. cause des mesures prises depuis 2018, le choix du niveau des dépenses locales a une moindre incidence sur la feuille d'impôt, sans compter que l'incitation à la bonne gestion a presque disparu. La solution ne réside pas dans un énième encadrement des finances des collectivités territoriales, comme le suggère la Cour. Elle repose au contraire sur la consécration- enfin ! -du couple libertés-responsabilités, autrement dit sur une autonomie accrue des élus locaux dans le cadre d'une décentralisation véritable qui ne serait plus une « coquille vide du groupe Union Centriste ne croient pas à la tutelle infantilisante de l'État. Au contraire, ils croient à la dialectique démocratiquement vertueuse des interactions entre électeurs, contribuables et usagers du service public. Une véritable décentralisation présenterait deux atouts majeurs. Elle conduirait à une gestion plus économe des ressources fiscales et à une structure des dépenses publiques s'accordant davantage avec les préférences politiques concitoyens. Une véritable décentralisation financière aurait des vertus cognitives que le centralisme jacobin n'a pas. Ce n'est Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le ratio des dépenses publiques par rapport au PIB est moins élevé dans les systèmes décentralisés que dans les systèmes centralisés, comme l'est le système français. La parole

de la croissance, qui a été rapide. Nous ne sommes pas des fourriers ou des parangons de l'austérité ; ce n'est absolument pas le cas.

de position fortes sur le rôle des communes. Je les partage, j'allais dire naturellement, puisque, dans une autre vie, j'ai moi-même été président d'un établissement public de coopération intercommunale. La réduction du nombre de communes

Monsieur Patient, le bilan de la décentralisation tel qu'il est dressé dans ce rapport public annuel ne traite en effet pas des collectivités d'outre-mer, parce qu'il nous a semblé que leur spécificité

au programme de la Cour. Je pense en outre que le rapport public annuel 2024 permettra de traiter de nombreux sujets les concernant ; nous nous engageons dans cette direction. Monsieur le sénateur Cozic,

le président de cette formation, le rapporteur général, moi-même, ou tel ou tel magistrat de la Cour, nous sommes naturellement à votre disposition. Je conclus mon propos en vous remerciant une nouvelle fois de votre participation à ce débat et de l'estime que vous avez témoignée aux travaux de la Cour. Je veux vous redire à quel point nous sommes

J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers